la commission des finances a émis un avis favorable- 35 voix pour, aucune voix contre et 3 bulletins blancs -à la reconduction de M. Nicolas Dufourcq aux fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.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 le groupe de travail dont les membres ont été nommés en séance le 17 janvier dernier, peut être transformé en commission spéciale. Il n'y a pas d'opposition ? ... Il en est ainsi décidé. demande du groupe Union Centriste, de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

« le besoin de s'aider engendre la bienveillance, une indulgence mutuelle, l'absence de toute rivalité », disait George Sand. Comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je crois en cette solidarité qui nourrit effectivement la bienveillance et contribue au changement de regard sur les plus fragiles. Elle renforce le lien social entre nos concitoyens et rappelle que les difficultés que peuvent rencontrer certaines familles à un moment donné sont l'affaire de tous et nous concernent tous, car nous sommes tous susceptibles de vivre un jour ou l'autre une épreuve de la vie qui nous fera apprécier cette solidarité que nous appelons de nos voeux. C'est cette solidarité qui nous rassemble aujourd'hui au travers de l'examen de cette proposition de loi loi visant à étendre le dispositif de don de jours de repos non pris aux aidants familiaux. L'enjeu est de taille, car ce sont 8 millions à 11 millions de Français, en grande majorité des femmes, qui aident régulièrement un de leurs proches en situation de handicap ou de dépendance, quel que soit leur âge. quel que soit leur âge. En tant que maman d'une enfant en situation de handicap, je connais bien le rôle essentiel des aidants, l'énergie, la force, le courage et le dévouement dont ils font preuve au quotidien, et je leur voue une grande admiration. Si nous travaillons tous dans le sens de la promotion d'une société inclusive, clef de voûte de ma feuille de route, nous devons pour autant faire preuve d'une grande vigilance, veiller à ce que l'inclusion ne se fasse pas au détriment de l'équilibre de vie des aidants et à ce que l'on ne fragilise davantage des familles déjà ébranlées. C'est pourquoi cette proposition de loi est particulièrement opportune. Le rôle des aidants va s'amplifier avec le temps. Vous savez, tout comme moi, que l'évolution démographique de notre pays constitue autant une chance qu'un défi. Nous avons besoin des aidants et nous devons les reconnaître, les soutenir, les préserver, car leur dévouement à un prix. Les aidants présentent d'ores et déjà 60 % de risques supplémentaires de contracter une maladie liée au stress et au surmenage. Rappelons-le, près de la moitié des aidants sont des actifs. Ils- et surtout elles, je le redis -doivent tout mener de front. Comme l'avait justement précisé la ministre du travail, Muriel Pénicaud, devant les députés, il existe une forte interaction entre la vie personnelle de l'aidant et son activité professionnelle. L'articulation entre ces vies constitue un défi quotidien qui le dépasse et affecte l'ensemble de son environnement professionnel, qui doit s'organiser d'une part pour pallier ses absences, d'autre part pour l'accompagner dans cette période difficile lorsqu'il est présent sur son poste de travail. Il s'agit là d'un enjeu majeur, sur lequel les employeurs, les ressources humaines, les partenaires sociaux doivent monter en puissance, en s'inspirant de pratiques volontaristes d'ores et déjà adoptées dans certaines entreprises. C'est donc en apportant la sécurité juridique nécessaire au mouvement de solidarité dans le monde du travail que nous soutiendrons et favoriserons la solidarité intergénérationnelle entre proches. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons la responsabilité collective de reconnaître ce rôle si exigeant des aidants en les soutenant dans leur engagement. Cette proposition de loi ne répond certes pas à l'ensemble des enjeux considérables relatifs à la situation des aidants familiaux, mais elle représente un pas significatif. Je veux rappeler à cet égard que j'ai confié, avec mes collègues Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, et Muriel Pénicaud, ministre du travail, une mission à Mme Dominique Gillot, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées et ancienne sénatrice. Son objet est de soutenir le retour et le maintien dans l'emploi des aidants familiaux de personnes en situation de handicap ou de personnes âgées. Dominique Gillot nous rendra en mars prochain ses conclusions. Elles pourront enrichir, le cas échéant, l'élaboration du projet de loi relatif à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Vous l'aurez compris, cette proposition de loi me tient à coeur. Le cap de la politique du handicap, dont le Président de la République a fait une priorité, est de faire de la France une société pleinement inclusive. Or une société inclusive ne peut se penser sans tous ces proches qui soutiennent et accompagnent les projets de vie du quotidien des personnes en situation de handicap et de dépendance. Le Gouvernement est mobilisé pour améliorer le soutien aux aidants, véritable gage d'une meilleure qualité du soutien présent et futur à nos personnes âgées et en situation de handicap. Pour toutes ces raisons, madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement donne un avis favorable à cette proposition de loi.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

millions selon certaines sources -à apporter leur aide, quotidienne et bénévole, à un membre de leur entourage proche. L'explosion de leur nombre est une conséquence directe de l'allongement de la durée de la vie et du désir qu'ont les personnes en perte d'autonomie de se maintenir chez elles : autant d'heureuses tendances dont on a trop longtemps négligé les effets. Tout à la joie de pouvoir jouir plus longuement de nos proches, nous oublions souvent que la fragilité qui accompagne l'âge ou le handicap exige que nous nous acquittions envers eux d'un surcroît de soins et d'attention. Mes chers collègues, les proches aidants, les aidants familiaux, ces personnes dont le droit n'a pas encore figé l'appellation, connaissent une détresse profonde. Sourde et digne, souvent inexprimée parce qu'issue d'un mouvement qu'animent indistinctement devoir et compassion

Quand la personne s'abîme doucement, quand sa carrière est compromise, quand sa propre famille se fissure à force de vivre deux vies, la sienne et celle dont elle s'est donné la charge, alors notre devoir ne se résume plus à laisser à la société le soin de réguler d'elle-même ses propres cellules d'apporter l'élément qui éveillera les consciences sur une réalité trop souvent ignorée. Cet élément, le voici. Il n'est certes pas parfait. Le mérite de ce texte revient à notre collègue député Paul Christophe, du groupe UDI, Agir et Indépendants, qui l'a inscrit à l'ordre du jour réservé aux groupes minoritaires de l'Assemblée nationale. Il constitue une transposition aux proches aidants du dispositif de la loi du 9 mai 2014, également issu d'une initiative parlementaire et visant à permettre aux collègues d'un salarié dont l'enfant est atteint d'une maladie grave

les petites et moyennes entreprises, où les jours de congés au-delà du seuil légal sont presque inexistants, la loi ne se distinguait guère d'une simple déclaration d'intention. Pourtant, le Parlement l'a votée, parce qu'il s'agissait d'une main tendue, parce que, malgré le risque de voir ses effets partiellement neutralisés, elle disait aux parents d'enfants gravement malades, avec la solennité dont la loi seule peut être revêtue, la considération, l'empathie et l'appui des pouvoirs publics. C'est ce geste que je vous demande de renouveler aujourd'hui. Je n'en partage pas moins l'insatisfaction de certains de mes collègues. Je suis tout à fait consciente que la discussion d'un nouveau texte sur les proches aidants de personnes âgées ou handicapées nous fait passer à côté de la réforme ambitieuse et d'envergure que leur condition réclame. Je suis tout à fait consciente que le don de jours de congés payés au proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ne répond que très imparfaitement aux besoins réels qu'une pareille situation implique

soit tenu, et surtout à ce qu'il intègre la condition des proches aidants de personnes âgées. Forts de cet engagement, je vous demande donc, mes chers collègues, de voter cette proposition de loi en l'état. Je vous demande de me rejoindre dans une patiente détermination à donner aux aidants les droits qui leur sont nécessaires, et à leur adresser pour l'heure le signal qu'ils ne sont pas oubliés et que la représentation nationale prend leurs intérêts à coeur. Songez bien que la modification de ce texte, inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale réservé aux groupes minoritaires, contraindrait nos assemblées à poursuivre une navette dont l'aboutissement demeure plus qu'incertain. Nous ne perdrions certes pas l'occasion d'inscrire un droit essentiel au côté de ceux qui existent déjà, mais nous passerions à côté de celle, dont il est rarement donné au Parlement de se saisir, d'adresser aux aidants un geste fort, que je veux riche de promesses. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement, longtemps attendu, de reconnaissance des aidants.

Les termes « aidant familial » ou « proche aidant » qui désignent ceux qui assurent cette forme exigeante de secours à un proche ne sont apparus que relativement récemment. Longtemps en effet ils- ou plutôt elles -ont été invisibles dans nos politiques publiques. le plus souvent épouses, mères ou filles des personnes qu'elles assistent, la spécificité de leur engagement, et donc de leurs besoins, a d'abord été ignorée, parce que relevant d'une solidarité familiale perçue comme naturelle, mais reposant pourtant de façon disproportionnée sur les femmes. Puis le regard porté sur les aidants a changé : collectivement, nous reconnaissons désormais leur apport spécifique à notre système de solidarité et avons pris conscience qu'il faut « aider les aidants Depuis plus de dix ans maintenant, comme vous le rappelez dans votre rapport, madame la rapporteur, plusieurs dispositions ont été adoptées pour reconnaître des droits sociaux aux aidants, notamment salariés, comme le droit à congé, à la retraite ou, dans certains cas, l'ouverture de possibilités de dédommagement.

En complément, la loi du 9 mai 2014, ou loi Mathys, a encouragé la solidarité horizontale en généralisant la possibilité de faire le don de jours de repos à un collègue pour lui permettre de rester auprès de son enfant gravement malade. Aujourd'hui, nous complétons ce dispositif en l'étendant au « salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap ». Cette extension concernera également la fonction publique. Certes, les quelques jours de repos ainsi collectés ne permettront pas aux aidants de faire face sur le long terme- souvent plusieurs années -aux difficultés liées à la perte d'autonomie de leur proche. pas en avant supplémentaire est bienvenu. Nous soutiendrons ce texte par notre vote unanime, car il participe du changement culturel qui s'opère dans notre société au bénéfice des aidants. Pour autant, nous devons constater l'émiettement des dispositions actuelles en faveur des aidants, ainsi qu'un manque de lisibilité du champ des personnes concernées et de leurs droits. Il y a donc urgence à définir une stratégie globale pour les aidants, notamment celles et ceux qui ont une activité professionnelle. On ne peut pas continuer ainsi à se pencher sur leur situation au coup par coup. En raison de l'allongement de la durée de la vie, du recul de l'âge de la retraite, du souhait de rester chez soi, du manque de structures et du coût de celles-ci, chacun, un jour ou l'autre, peut être amené à devenir aidant d'une personne en perte d'autonomie tout en ayant une activité professionnelle,

leur proche sont multiples : nécessité de réduire ses horaires de travail, absences fréquentes, choix d'un métier ou d'un poste moins rémunérateur mais moins contraignant, refus de promotions, fatigue, voire épuisement, qui affecte la productivité au travail, et malheureusement, dans certains cas, hostilité, voire discrimination. L'enjeu de société est doublement important, car de 60 % à 70 % des aidants sont des femmes, qui souffrent déjà des inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Pour réduire ces inégalités, toutes les solutions doivent être mobilisées : renforcement de l'accès géographique et économique aux services d'aides à domicile pour soulager les aidantes avec les entreprises, sur l'aménagement du temps de travail et le recours au télétravail lorsque c'est pertinent. L'aidant ne doit pas être perçu négativement dans la collectivité de travail. Il faudra également développer les mécanismes de solidarité collective pour compenser les pertes de revenus et de cotisations résultant des réductions ou interruptions temporaires d'activité. Le vote d'aujourd'hui n'épuisera donc pas, tant s'en faut, la question du soutien aux aidants, mais il sera le gage de notre mobilisation.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord de remercier Mme la rapporteur de la qualité et de l'objectivité de son rapport. Nous apprécions particulièrement, au groupe communiste républicain citoyen et écologiste, qu'elle n'ait pas caché les limites de cette proposition de loi. Pour nous aussi, la générosité est une valeur que la société doit savoir promouvoir. Notre réticence à l'égard de ce texte ne se situe donc pas à ce niveau. Permettre à des salariés de faire don de jours de congés au-delà de la durée légale, pourquoi pas ?

Mais surtout, comme l'a d'ailleurs rappelé la présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, « il revient aussi à la solidarité, aux politiques publiques de financer l'effort nécessaire nous dirions même qu'il revient à l'État de donner l'exemple. Or vous soulignez vous-même, madame la rapporteur, que « cette proposition de loi ne saurait en aucun cas prétendre corriger toutes les carences très importantes dont les droits de l'aidant continuent aujourd'hui de souffrir », et vous donnez rendez-vous au Gouvernement sur ce sujet. Nous proposons, là encore, d'aller plus loin. Tel est le sens de l'amendement de fond que nous avons

Notre collègue député Pierre Dharréville vient de dévoiler toute une série de propositions en conclusion de la « mission flash » qu'il a menée sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Tout d'abord, pour promouvoir le recours au congé de faible, il propose de créer une indemnisation dont le montant pourrait être identique à celui de l'allocation journalière de présence parentale, soit 43,14 euros par jour.

Ensuite, les proches aidants de personnes handicapées bénéficiant déjà d'une majoration de leur durée de cotisation à l'assurance vieillesse, à hauteur d'un trimestre par période de prise en charge de trente mois, dans la limite de huit trimestres, collègue député propose d'étendre ce système pour en faire bénéficier aussi les proches aidants de personnes âgées dépendantes. Enfin, il est proposé de prendre en charge à 100 % les dépenses de santé des aidants, en raison de leur état d'épuisement physique et mental, qui nécessiterait

Nous entendons votre argument, mais si nous votions ce texte en l'état, nous dédouanerions encore une fois le Gouvernement de ses obligations ! Quant à la nécessité d'aller vite, faut-il rappeler qu'il a fallu attendre près d'un an les décrets d'application de la loi du 9 mai 2014 relative aux enfants malades

un accident de voiture, l'annonce d'une maladie auto-immune, des parents dont il faut s'occuper dans l'urgence : on ne s'y attend pas, on est dans le feu de l'action, on exerce son activité professionnelle, on jouit de la sérénité familiale, mais la vie bascule. Il faut faire face ! La famille, les proches doivent affronter avec courage une situation qui exigera non seulement de la force morale et psychologique, de la résistance physique, mais aussi une capacité financière certaine. Nous payons bien souvent les carences de l'État. Il faut opérer des sacrifices professionnels, personnels, mais la réaction s'organise et se structure. La vie est la plus forte, et il faut aller de l'avant pour accompagner des personnes fragilisées et devenues dépendantes. Hier, la question ne se posait pas. Nos vieux parents étaient accueillis dans le creuset familial. Nous gardions, devant le handicap, un silence pudique. C'était une « affaire de famille », presque secrète. Puis, peu à peu, les langues se délient, les témoignages se déploient, les demandes de soutien se précisent : on en parle ! De nouveaux phénomènes interpellent la société, comme la découverte de certaines maladies ou, plus heureusement, l'allongement de la durée de vie.

rappelées dans les rapports de Paul Christophe, député des Flandres, et de notre collègue rapporteur, Jocelyne Guidez -qui ont conduit à la création du statut d'aidant familial. Cette expression est la transposition d'un vocable technocratique. Elle devrait refléter le seul élan du coeur, la simple générosité, mais le législateur n'est pas un poète ! Il doit qualifier juridiquement des situations humaines. Il faut donc aider les aidants.

L'objet de cette proposition de loi est simple, mais louable : étendre le dispositif du don de jours de repos aux salariés confrontés à la nécessité de s'occuper d'une personne qui n'est plus autonome.

dans l'introduction de son excellent rapport de stage de 2007, intitulé « Enquête auprès des aidants familiaux des personnes âgées en perte d'autonomie », Mohamadou Oumarou Danni, alors étudiant de master 2 à l'université de Poitiers, faisait état d'une situation qui, plus d'une : « Le vieillissement progressif de la population française et l'accroissement de la dépendance physique et psychologique qui en résulte constituent un phénomène lourd que toutes les projections démographiques confirment. Ainsi, la société française, comme la plupart des sociétés occidentales, est et va être durablement affectée par cette situation qui, directement ou indirectement, concernera à moyen ou à long terme toutes les familles. Cette augmentation du nombre de personnes en situation de handicap pose évidemment la question de leur prise en charge, car il n'existe pas assez de places en maisons de retraite ou en établissements spécialisés pour les accueillir. Pour faire face à ce défi majeur, les pouvoirs publics privilégient de plus en plus le maintien à domicile, mais, pour ce faire, il semble nécessaire, voire primordial, de créer un environnement favorable aux conditions de travail d'aidant. » d'aidant. » Mes chers collègues, vous le voyez, onze ans plus tard, la problématique reste d'actualité. Il faut bien l'admettre : malgré la qualité de notre système de soins et de santé, les progrès de la médecine, le matériel innovant toujours plus moderne et plus efficace, il n'est toujours pas possible d'assurer entièrement une bonne prise en charge des personnes en situation de handicap. Les proches aidants jouent donc un rôle fondamental, et l'État ne peut entièrement se substituer comme le soulignait Mohamadou Oumarou Danni, c'est justice de donner davantage de moyens aux proches aidants pour assumer ces tâches quotidiennes qui viennent s'ajouter à celles des vies familiale, professionnelle et personnelle.

loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, enfin à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans cette lignée, en tendant à permettre à un salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise étant un proche aidant et à condition de conserver un minimum de vingt-quatre jours de repos, conformément au droit européen. On ne peut que saluer ce dispositif, qui va dans le bon sens, même s'il n'est pas parfait. Ainsi, il faudra probablement décliner l'applicabilité de ce texte selon la taille des entreprises. De leur côté, ces dernières devront faire preuve de la plus grande souplesse pour adapter au mieux, selon leurs moyens et leurs possibilités, les présentes dispositions.

eux-mêmes. Pour bon nombre de nos concitoyens, il est difficile de trouver un équilibre entre travail et vie privée. Imaginez la situation dans laquelle se trouvent ceux qui, parmi nous, doivent également assumer la charge d'une ou de plusieurs personnes en perte d'autonomie

Je tiens à saluer ce travail, sa pertinence et la profondeur de la réflexion conduite. Mes chers collègues, les élus du groupe du RDSE ont, à l'unanimité, choisi de se conformer à la demande de Mme la rapporteur de ne pas amender le texte afin que son adoption par le Parlement- et donc son entrée en application -puisse

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté aujourd'hui a fait l'objet d'un large consensus à l'Assemblée nationale. Nul doute qu'il en ira de même au Sénat. Je suis particulièrement heureux d'intervenir dans cette discussion générale. En effet, cette proposition de loi visant à étendre le dispositif de dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux s'inspire assez largement de la loi du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, soutenue par M. Paul Salen, député de la Loire qui, à l'époque, était également mon premier vice-président au conseil départemental. avait eu connaissance de la détresse et des difficultés des parents d'un enfant atteint d'un cancer en phase terminale. Ces parents voulaient, bien entendu, rester près de leur enfant et l'accompagner le plus possible dans cette terrible épreuve. M. Salen avait-il proposé ce dispositif afin de répondre à des situations ponctuelles d'urgence. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a pour objet d'encourager, par une sécurisation juridique accrue, les élans de solidarité entre collègues de travail lorsque l'un d'eux traverse une période particulièrement difficile du fait du poids de son rôle auprès d'un proche en situation de handicap ou auprès d'une personne âgée en perte d'autonomie. Toutes les études le démontrent : les aidants, souvent issus de la fameuse « génération pivot », représentent la solution d'accompagnement privilégiée par les personnes concernées par la perte d'autonomie d'un proche. C'est aussi la solution la moins coûteuse, loin devant les aides professionnelles à domicile et l'accueil La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a permis des avancées majeures au bénéfice des aidants familiaux, en reconnaissant leur engagement au travers de la définition du statut de « proche aidant qui va bien au-delà des seuls membres de la famille. Ce texte a aussi introduit plusieurs dispositifs visant à accompagner, à informer et à former les aidants, ainsi qu'à mieux prendre en compte leurs besoins, en créant le congé de proche aidant et le droit au répit. il est clair que la santé des aidants est un enjeu de santé publique. Il faudra veiller à ce que les dispositifs prévus dans les textes précités soient efficacement mis en oeuvre. Plusieurs missions en cours devraient nous éclairer sur ce point.

Il a le mérite de permettre un aménagement et un allégement du temps de travail des aidants familiaux sans que ces derniers aient à subir une perte de salaire. Pour autant, si elle part d'une intention tout à fait louable et respectable, à laquelle, bien sûr, je souscris, cette proposition de loi ne répond pas totalement totalement à un certain nombre de difficultés que pourraient poser ses modalités d'application et de mise en oeuvre. Permettez-moi de m'arrêter sur certaines d'entre elles. Premièrement, le don concerne les jours de repos excédant les vingt-quatre jours de congés payés annuels.

Comment des salariés pourront-ils aider un collègue sur une très longue période ? Quelle peut être l'incidence de ce soutien, non seulement en termes financiers, mais aussi sur le fonctionnement de l'entreprise ? Troisièmement, quelles seront les conditions d'application de ce dispositif dans la fonction publique ? Quatrièmement, le présent texte ne prend pas en compte la situation de celles et ceux qui ont dû abandonner leur travail pour s'occuper de personnes âgées dépendantes. À quand une harmonisation de leurs droits avec ceux des proches aidants des personnes présentant un handicap ? Plus généralement, ne faudrait-il pas réserver cette faculté de bénéficier d'un don de jours de repos à des salariés se trouvant brusquement en situation d'urgence et ayant ponctuellement besoin de se rendre disponibles pour faire face à un accident de la vie, sans qu'il s'agisse obligatoirement d'aider des personnes âgées ou handicapées ?

pourrait aussi, de manière induite, nous permettre de renforcer les liens intergénérationnels au sein des familles, dans la mesure où ce sont bien souvent les enfants qui prennent en charge leurs parents âgés ou dépendants.

cette proposition de loi relative au don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants, il s'agit de faire face à des situations de crise conjoncturelles pour les aidants, dont l'implication psychologique est déjà très forte tout au long de l'année.

On parle aussi souvent d'aidant informel, c'est-à-dire non professionnel, venant en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie. parler d'aidants, c'est bien parler de la vie de tous les jours : une fin de vie, une maladie, un cas d'Alzheimer identifié, une tumeur suspectée, la naissance d'un enfant différent, et nous devenons tous des aidants naturels.

Ensuite, vous avez fait preuve d'un certain courage en préconisant l'adoption conforme de cette proposition de loi, afin d'en assurer la promulgation rapide. et de responsabilité, car il y aurait tant à faire ! Mes collègues ont déjà donné quelques pistes. Vous avez raison d'appeler à une réflexion d'ensemble sur la question des proches aidants, qui ne fait l'objet que de mesures parcellaires disséminées dans plusieurs textes de loi. La première véritable prise en charge de la

matière, il existe également des accords d'entreprise. Quelle est la plus-value du texte que nous examinons aujourd'hui ? Il complète la loi du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade. Le cadre juridique est strictement repris et élargi aux personnes prenant en charge

si le dispositif proposé peut permettre, dans des situations exceptionnelles, à des élans de générosité de s'exprimer librement, il n'assure pas la reconnaissance du statut juridique du proche aidant.

Centriste pensent qu'il est nécessaire de travailler à une approche plus globale. Les proches aidants ont besoin de moyens, de temps, de compensations et de reconnaissance.

les aidants sont souvent les conjoints des personnes dépendantes, mais ce sont aussi les enfants, les petits-enfants ou des membres de la famille qui prennent sur leur temps pour accompagner la personne en perte d'autonomie, que ce soit en raison d'une maladie, d'un handicap ou du vieillissement. Selon la

toutes les zones n'étant pas pourvues d'établissements spécialisés. Si la solidarité familiale et le rôle social des aidants sont réels, notamment en milieu rural, ils masquent difficilement les carences de la société en matière de prise en charge.

Le don de jours de congé aux proches aidants, transposition du dispositif de la loi Salen, est incontestablement une réponse à prendre en compte. L'ouverture de ce droit légitime est d'ailleurs très attendue par les familles, et nous y sommes très favorables.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur, mes chers collègues, comme l'a indiqué Jean-Pierre Decool, cette proposition de loi complète les avancées de la loi Paul Salen, qui a permis le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade. Elle étend ce dispositif de don de jours de repos à tous les aidants, quel que soit l'âge de la personne dépendante. Dans le cadre du maintien à domicile, les personnes âgées et les personnes handicapées ont un projet de vie financé par l'APA ou

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a pour objet de créer un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants. Je tiens à saluer cette initiative et, plus largement, le travail de nos collègues de l'Assemblée nationale : par voie d'amendement, ils ont élargi le champ d'application de ce dispositif aux proches aidants de personnes présentant un handicap.

En effet, certaines familles ne peuvent bénéficier rapidement de réponses adaptées à la situation de la personne qu'elles accompagnent, ce qui leur impose d'assurer une présence à domicile. Parfois, il s'agit d'un choix délibéré de la famille, fait pour le bien-être de la personne

Je citerai notamment la loi de 9 mai 2014, chère à notre collègue Bernard Bonne, qui permet à un salarié de donner des jours de repos à un collègue dont l'enfant est gravement malade, la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, qui donne une définition légale du proche aidant et lui permet l'accès aux dispositifs du congé de proche aidant et du droit au répit, la loi du 8 août 2016, dite loi El Khomri, qui accorde aux parents d'enfant handicapé deux jours de congé supplémentaires par an. nous ne pourrons pas faire l'économie d'un texte tendant à définir un véritable statut de l'aidant et prenant en compte toutes les situations, qu'il s'agisse des personnes handicapées, en perte d'autonomie, gravement malades ou en fin de vie. Comme vous l'avez dit, madame la secrétaire d'État, nous devons être conscients que ces situations se répercutent sur la vie professionnelle, familiale et personnelle des aidants. Le Parlement doit être force de proposition et se saisir de ce sujet,

Pourquoi ne pas imaginer la création d'un congé parental spécifique, notamment pour les parents aidants d'enfants handicapés, pour lesquels il n'existe pas de prise en charge, ou d'enfants en longue maladie ? Les droits sociaux des aidants à la retraite ou au chômage représentent également des enjeux importants, de même que la reconversion professionnelle.

Concernant le coût de ces nouvelles mesures, n'oublions pas que l'inclusion dans le milieu ordinaire, le maintien d'une personne à domicile, lorsque cela est possible, sont moins coûteux que la création de places, de chambres dans les institutions.

Watrin. Comme je l'ai indiqué lors de la discussion générale, cet amendement d'appel vise à obtenir du Gouvernement des engagements précis sur la mise en place de mesures concrètes en faveur des aidants. Nous refusons de faire reposer sur la seule générosité des salariés l'accompagnement, ô combien nécessaire, des proches aidants qui s'occupent des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Il est de la responsabilité collective des pouvoirs publics de prendre des dispositions non seulement nécessaires, mais aussi attendues.

hauteur du montant actuel de l'allocation journalière de présence parentale. L'absence d'indemnisation est un obstacle souvent rédhibitoire à la mobilisation de ce congé. Nous proposons, ensuite, d'étendre la majoration de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse dont bénéficient les personnes handicapées aux proches aidants. Une majoration d'un trimestre par période de prise en charge de trente mois, dans la limite de huit trimestres, représenterait une avancée dans la compensation de l'investissement des proches aidants sur le plan de la retraite. Nous proposons, enfin,

même, mon cher collègue ! Votre amendement illustre parfaitement le dilemme que j'ai évoqué lors de la discussion générale. Je partage sans réserve les préconisations de notre collègue député Pierre Dharréville, et je suis favorable à ce que les droits sociaux des proches aidants soient homogénéisés et renforcés.

Au surplus, les mesures pour lesquelles vous demandez une évaluation par le Gouvernement font l'objet d'une proposition de loi déposée par M. le député Pierre Dharréville, qui sera discutée à l'Assemblée nationale le 8 mars prochain,

conduisant souvent certains et certaines à mettre de côté leur vie professionnelle, voire leur vie personnelle. Ce rôle d'aidant familial est souvent vécu comme une charge lourde, tant sur le plan psychique que sur les plans physique, émotionnel, social et financier. Le présent texte, même s'il ne résout pas tout, est très attendu par les quelque 8,3 millions d'aidants en France, dont 18 000 en Martinique, qui prennent soin d'un proche dépendant, malade ou handicapé.

Le groupe Les Indépendants-République et Territoires se félicite de l'accueil réservé à cette proposition de loi du député Paul Christophe, qui traduit un bel élan d'unanimité de la classe politique, dépassant les clivages partisans. La

de plus de 65 ans ; ils seront 20 millions en 2030 et 24 millions en 2060. Nous sommes donc la première génération à en assumer d'autres : celles de nos enfants et de nos petits-enfants, la nôtre et, souvent, celle de nos parents ... Nous n'avons pas le choix, il est de notre devoir d'anticiper en donnant un cadre juridique à ces initiatives spontanées. Certes, nous avons conscience des insuffisances des dispositifs, mais nous tentons de répondre à des situations concrètes.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que le représentant du groupe auteur de la demande disposera d'un temps de parole de dix minutes,

Symbole emblématique de liberté, d'aventure et d'indépendance, la voiture tend à devenir une réelle contrainte pour les personnes vivant en milieu urbain, alors qu'elle reste indispensable en milieu rural.

Avec l'apparition des nouvelles formes de mobilité, cet objet de convoitise tend à devenir un moyen de transport contraignant. Plus étonnant, c'est la voiture qui semble vouloir s'émanciper et reprendre sa liberté, puisqu'elle va probablement bientôt pouvoir se passer de conductrice ou de conducteur. Le véhicule autonome est présenté comme le moyen radical de réduire la mortalité sur les routes, surtout dans des pays comme les États-Unis, où la mortalité routière atteint des taux record, deux fois supérieurs à ceux que l'on observe en Europe. On attend beaucoup du véhicule autonome, en espérant qu'il permettra de se déplacer partout avec facilité, à un coût maîtrisé. La France a une carte à jouer dans ce domaine, malgré un retard à l'allumage que l'on ne peut pas nier.

mais aussi une vingtaine d'industriels, dont certains implantés à Toulouse, comme Continental ou Renault avec ses Software Labs. Vous avez récemment eu l'occasion, madame la ministre, d'expérimenter la navette autonome développée par la start-up Easymile sur l'ancien aérodrome de Francazal. Les constructeurs Renault et PSA, tout juste sortis d'une crise difficile, tentent de prendre pied sur le marché de la voiture autonome. La concurrence est rude, elle dispose d'énormes moyens et va très vite. concerne les équipementiers, Valeo semble tout à fait au niveau, mais, à l'ère du numérique, les retournements peuvent se produire à la vitesse de l'éclair. Le robot-voiture, conçu comme un salon sur roues assumant la totalité du trajet, quels que soient l'état de la route ou les conditions météorologiques, reste une perspective de long terme.

Les espoirs sont également réels en matière de protection de l'environnement, nos véhicules thermiques étant devenus indésirables dans les grandes villes, pour des raisons évidentes de qualité de l'air et de santé publique.

Tous les responsables politiques ont bien compris que nous étions parvenus au bout d'un système. Il faut absolument sortir les véhicules thermiques des grandes agglomérations telles que Paris, Lyon, Toulouse ou Marseille. Ce sera possible si les élus responsables peuvent proposer des solutions alternatives. Le véhicule ou la navette autonome semble ouvrir une nouvelle voie en matière de circulation urbaine et offrir une réelle perspective de substitution aux véhicules thermiques, devenus indésirables en ville. Il représente une solution démocratique pour assurer les transports de tous les citoyens dans les grands centres urbains. C'est certainement la révolution de demain ! Ces navettes autonomes viendraient compléter les transports existants, comme le tram ou le métro, en irriguant les plus petites artères. Depuis quelque temps, les aides à la conduite ont déjà fait leur apparition dans certains véhicules : régulation de vitesse adaptative, stationnement accompagné, système de lecture des panneaux et d'évitement des obstacles. Aujourd'hui, la conduite sans chauffeur, qui commence à se développer dans des pays tels que les États-Unis, la Chine et le Japon, soulève des questions auxquelles il sera nécessaire d'apporter rapidement des réponses concrètes afin de ne pas se laisser dépasser dans le domaine des technologies de demain. demain. La route est longue, et commence par une évolution des mentalités. Les clients ne semblent pas tout à fait prêts. Selon le baromètre annuel 2016 aramisauto.com/TNS Sofres % de nos concitoyens appréhendent un manque de fiabilité de ces véhicules et redoutent de lâcher le volant. Ils sont même 75 % à craindre de perdre le plaisir de conduire. Au vu de la diversité des enjeux liés à la voiture autonome, force est de constater que les défis sécuritaires, économiques, technologiques, éthiques et réglementaires à relever pour faire de ce mode de transport une réalité véhicule autonome et connecté requiert des avancées non négligeables en termes d'infrastructures routières afin d'accompagner l'acquisition et le traitement des images. Il nécessite une harmonisation technique entre véhicules et véhicules ainsi qu'entre véhicules et infrastructures. À ce jour, il n'existe pas de chiffrage précis des investissements nécessaires, mais il est indispensable de traiter le sujet du financement de l'adaptation des infrastructures routières à la conduite sans chauffeur. En préalable au développement il faut réaliser des investissements gigantesques pour moderniser les voies de circulation. Sur le plan juridique, alors que de nombreux pays avancent de manière significative- les États-Unis ont pris une avance déterminante en permettant à titre expérimental, depuis septembre dernier, la circulation de 100 000 véhicules sur toutes les voies -, il est urgent que l'Union européenne fasse juridiquement le choix de l'intelligence artificielle et tranche les choix moraux qui s'y rapportent. L'impossibilité d'opérer au sein d'un même cadre juridique est un obstacle majeur pour l'Union européenne. L'Europe et les États-Unis ont retenu deux approches différentes en ce qui concerne la réglementation des véhicules autonomes. L'Europe suit la ligne de conduite qui est la sienne depuis l'origine en matière de réglementation, le principe de base étant la fourniture d'un cadre réglementaire complet aux entreprises qui souhaitent développer cette technologie afin qu'elles puissent adapter leurs véhicules en conséquence. Elles auront alors l'assurance, si elles respectent scrupuleusement les réglementations en vigueur, de ne pas être poursuivies en cas d'incident ou d'accident. Les États membres de l'Union européenne cherchent à faire évoluer les réglementations existantes et à en adopter de nouvelles pour sécuriser la situation des véhicules autonomes et leur fournir un cadre stable. Ainsi, la convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière, qui disposait que « tout véhicule en mouvement [ ...] doit avoir un conducteur a été amendée en mars 2016 afin d'autoriser explicitement les systèmes de conduite automatisée, comme sur les bateaux et les avions, à condition qu'ils soient conformes aux réglementations des États ou qu'ils puissent être contrôlés, voire désactivés, par le conducteur. Il demeure pourtant que, actuellement, un véhicule complètement autonome ne peut pas circuler dans les États membres de l'Union européenne, signataires de cette convention. Les États-Unis, eux, sont avantagés dans cette compétition par leur système plus permissif, qui autorise les constructeurs à poursuivre leurs expérimentations dans un nouvel État quand un autre les interdit. En France, le processus d'expérimentation est bien plus lourd qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne, et nous avons quelques mois de retard sur nos homologues européens en matière de textes réglementaires. Les constructeurs allemands ont fait pression sur leurs autorités pour que les fonctionnalités d'autonomie qu'ils souhaitaient installer sur leurs véhicules fassent l'objet d'une dérogation à la convention de Vienne. Les constructeurs français souffrent d'un manque de souplesse et pourraient être amenés à en pâtir de nouveau dans le futur. En outre, la responsabilité des robots, la protection des données individuelles soulèvent des difficultés que nous avons également du mal à surmonter. Les pays européens s'interrogent sur la détermination de la responsabilité en cas d'accident. En effet, la conduite sans chauffeur introduit de nouvelles parties à la chaîne des responsabilités. Il s'avère aujourd'hui nécessaire de définir les règles applicables au développement de la robotique et d'établir les responsabilités de chacun dans ce processus. De plus, permettre à un ordinateur de gérer l'intégralité de la conduite d'un véhicule rend indispensable la mise en place de systèmes de cybersécurité ultraperformants pour éviter la prise de contrôle des véhicules autonomes par un tiers malveillant. Au vu des nombreuses problématiques soulevées par la conduite sans chauffeur, deux conclusions s'imposent sur le plan purement routier. Aujourd'hui, tandis que se développent très rapidement les aides à la conduite de véhicules de plus en plus assistés, il est nécessaire que les États membres de l'Union européenne harmonisent leurs positions dans les enceintes internationales afin que nos industriels puissent participer activement à cette révolution mondiale de la voiture autonome et réaliser des essais à grande échelle sur le vieux continent.

Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis très heureuse d'avoir l'occasion de débattre avec vous sur le sujet du véhicule autonome. L'arrivée des véhicules autonomes est un enjeu de société important. Le véhicule autonome va transformer notre manière de nous déplacer, notre rapport à la mobilité, nos filières économiques. Il nous faut préparer ces mutations en offrant un cadre favorable à l'innovation et protecteur, afin que la sécurité, dans toutes ses acceptions, soit assurée.

La conduite automatisée sur routes séparées est testée en conditions réelles. Les applications à la logistique urbaine voient le jour. D'autres modes de transport, notamment maritime, développent des solutions de conduite autonome. C'est le bon moment pour échanger, car le Gouvernement prévoit d'adapter, au travers du projet de loi d'orientation des mobilités que je construis et dont nous aurons à débattre d'ici à l'été, notre cadre à cette réalité, après avoir consulté l'ensemble des parties prenantes.

On sait que les facteurs humains, qu'il s'agisse de la consommation d'alcool, de la somnolence ou de la vitesse excessive, sont les principales causes d'accidents de la route. La délégation de conduite permettra de limiter l'impact de ces facteurs. Le second enjeu est celui de la qualité des services de mobilité. La voiture autonome apportera un confort accru lors des déplacements, mais c'est surtout en matière de mobilité partagée que l'on peut anticiper un apport décisif pour les Français, grâce notamment à de nouveaux services susceptibles de compléter l'ossature des transports en commun, rabattement ou un complément de desserte en période creuse ou en zones périurbaines ou rurales. Le troisième enjeu est celui de l'impact environnemental. Le véhicule automatisé devrait permettre une fluidification du trafic routier et un accroissement considérable de l'efficacité des mesures de régulation dynamique du trafic. Cependant, il réduira aussi le coût d'usage du véhicule motorisé et doit donc être propre

Des recompositions de la chaîne de valeur dans ces industries sont à prévoir, avec l'arrivée de nouveaux entrants. La France dispose d'atouts majeurs dans ce domaine, et c'est le rôle de la puissance publique

Médevielle, cette acceptabilité ne doit pas être considérée comme acquise. Il importe de mieux connaître les perceptions et les freins d'acceptabilité ou éthiques suscités par l'apparition du véhicule autonome. Comment la puissance publique- l'État, mais aussi les collectivités territoriales -peut-elle apporter une réponse face à ces enjeux ? La révolution du véhicule automatisé représente une opportunité majeure pour développer de nouveaux services, en milieu urbain comme en milieu rural,

Pour ces raisons, notre action devra être ambitieuse, déterminée et progressive. Mon ambition, celle du Gouvernement, est d'abord de construire un cadre légal et réglementaire qui permettra la circulation en toute sécurité des véhicules automatisés de série avant la fin du quinquennat. Cette ambition s'appuiera sur la mise en place d'un cadre d'expérimentation compétitif en cohérence avec le rythme de déploiement anticipé par nos filières. La progressivité est essentielle. L'élaboration du cadre réglementaire se fondera sur l'analyse des impacts et des risques identifiés lors des travaux menés en coopération étroite entre autorités publiques et industriels. Ces travaux devront permettre de construire le corpus de connaissances permettant l'évaluation et la validation des systèmes d'automatisation. Ce cadre totalement nouveau bouleversera la manière dont nous concevons la relation entre l'usage et le véhicule. Quelle forme prendra le permis de conduire de demain ? Comment l'usager doit-il être informé des capacités de son véhicule ?

Gérard Collomb, Bruno Le Maire, Mounir Mahjoubi et moi-même avons ainsi souhaité que l'État dresse un cadre d'action clair et ambitieux. C'est pourquoi nous avons nommé Anne-Marie Idrac haute responsable pour la stratégie nationale du développement des véhicules autonomes. Après avoir consulté constructeurs, acteurs du numérique, collectivités territoriales, usagers, opérateurs de transport de voyageurs et de marchandises et gestionnaires d'infrastructures, Anne-Marie Idrac a construit ce cadre d'action. Il sera finalisé dans les toutes prochaines semaines. Il répondra aux enjeux que j'ai évoqués et comportera notamment un programme d'expérimentation permettant de construire des outils d'homologation et d'évaluer les impacts sur les usages et l'acceptabilité.

La France va se doter d'un cadre d'action national, mais la compétition est mondiale, notamment avec les États-Unis et la Chine, pour ne citer que ces deux États. L'échelle pertinente est donc naturellement celle de l'Union européenne, qui doit être à l'avant-garde des innovations de rupture, comme le Président de la République le souhaite. La Commission européenne proposera une feuille de route en mai prochain. Notre cadre d'action alimente la préparation de ces travaux. De notre point de vue, il y a trois priorités. le financement. Le déploiement des véhicules autonomes et des infrastructures associées aura un coût important. La capacité de l'Union européenne à contribuer à cet effort sera déterminante, notamment au moment des débats sur le cadre financier post-2020. La deuxième Les règles de conduite sont encadrées par les conventions de Genève et de Vienne, auxquelles nous sommes parties. Nous travaillons activement à modifier ces textes afin qu'ils prennent en compte les évolutions engendrées par l'arrivée des véhicules autonomes, notamment en termes de responsabilité. Mais cela prend du temps, et sans attendre nous invitons l'Union européenne à réfléchir à l'opportunité de mettre en place un cadre réglementaire commun, de nature d'ailleurs à éviter des disparités au sein du marché intérieur. est l'interopérabilité. Il est indispensable qu'un véhicule autonome puisse franchir le Rhin, les Pyrénées ou toute frontière au sein de l'Union européenne. Nous avons d'ores et déjà travaillé avec l'Allemagne et le Luxembourg à la mise en place d'un site-test à nos frontières,

La voiture autonome constitue une révolution dans l'usage des transports. Aujourd'hui, l'autonomie est partielle. Elle devrait devenir totale après 2020. Si, de prime abord, cette innovation a pour objectif d'améliorer la sécurité, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la pollution locale et les problèmes de santé qui l'accompagnent, quelle sera cependant la place de l'humain ? Il est très difficile aujourd'hui de voir où l'État place le curseur entre encouragement de l'innovation et de la recherche et réglementation, face à des plateformes dont le pouvoir menace les États et bouleverse en profondeur l'organisation du travail, voire l'emploi. aujourd'hui, les géants du numérique sont en concurrence féroce avec les constructeurs automobiles. Ainsi, en 2015, on pouvait lire que la mise à disposition de voitures autonomes en autopartage, annoncée par Google, pourrait fragiliser durablement la filière automobile. Ce serait la remise en cause de nombreux emplois en France et en Europe, au niveau des réseaux de distribution, des réparateurs, des auto-écoles, voire des assurances, sans parler des menaces qui pèsent sur la protection des données personnelles. personnelles. Les membres du groupe CRCE ont toujours estimé que les données devaient être considérées comme un bien public, et non comme un simple instrument de profit. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu l'et les « communs » de données. À cet égard, il n'est pas anodin que Google ait annoncé qu'il ne construirait pas de véhicule, mais compte commercialiser des logiciels de conduite autonome, sachant que ces logiciels prendront une place toujours plus importante dans la valeur ajoutée du véhicule. du véhicule. Nous pensons qu'il est essentiel que le Parlement soit informé de manière plus suivie de l'état d'avancement des réflexions des différents groupes de travail qui ont été mis en place après le vote de la loi de transition énergétique,

technologique majeure et de créer les conditions pour qu'elle soit créatrice d'emplois, notamment en préparant les conversions nécessaires. Ces enjeux sont vraiment au coeur de la réflexion qui a été engagée par le Conseil national de l'industrie. je l'ai dit précédemment, 500 000 emplois dans la filière automobile et 700 000 emplois dans le transport routier de voyageurs et de marchandises sont concernés. Nous allons probablement assister à des transferts

d'identifier les impacts sur les filières et de nous proposer des plans d'action en termes d'évolution des compétences. Sur la base de ce premier rapport, qui sera remis au premier semestre, il nous faudra travailler avec le monde éducatif et les systèmes de formation pour nous assurer que nous anticipons bien les évolutions. D'ores et déjà, on peut saluer les réflexions engagées par les opérateurs de transports publics réunis au sein de la « nouvelle France industrielle » sur les nouvelles compétences liées à la supervision et à l'accompagnement des navettes automatisées.

J'imagine demain le véhicule autonome compléter un maillage ou offrir de nouvelles solutions de mobilité en zone rurale comme en milieu urbain. En ville,

Vous oeuvrez avec votre ministère de tutelle pour organiser la transition énergétique, pour réduire la part du nucléaire dans la production électrique française et augmenter celle des énergies renouvelables.

En tout état de cause, le fait de recourir à des véhicules électriques et de vouloir réduire la part du nucléaire ne nous amènera pas à mobiliser plus d'énergiescarbonées, le nucléaire ayant vocation à être remplacé par des énergies renouvelables.

représente un enjeu économique très important et nous attendons beaucoup de l'État en termes de structuration d'une filière industrielle qui, en Maine-et-Loire, est déjà bien implantée, avec l'équipementier Valeo ou Scania, très présent sur le segment des transports collectifs. La montée en puissance de cette nouvelle technologie pose également de nombreuses questions en matière d'aménagement du territoire. Les véhicules autonomes sont en effet hyperconnectés et leur fonctionnement nécessitera un accès sans défaillance aux réseaux numériques fixes et mobiles.

la couverture numérique apparaît donc comme un préalable à la mise en place de cette nouvelle mobilité individuelle ou collective. Il ne faudrait pas que les territoires peu denses en soient exclus. Cela reviendrait à renforcer les fractures numérique et territoriale ressenties par nos concitoyens, alors que les bouleversements technologiques actuels contribuent précisément à désenclaver nos territoires en leur permettant de saisir de nouvelles opportunités de développement économique. La 5G, qui est encore loin d'être une réalité pour nos concitoyens, apparaît comme la « technologie clé » pour le développement à grande échelle des véhicules autonomes. Par ailleurs, au-delà de l'accès au numérique, il est également nécessaire de se pencher sur la question des infrastructures routières, qui permettront le fonctionnement sécurisé des véhicules autonomes. Madame la ministre, pourriez-vous nous apporter des précisions sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour favoriser un développement équilibré et sécurisé de cette nouvelle technologie ? La parole

Les orientations nationales sur les cas d'usage et les impacts à évaluer prioritairementdonnent toute leur place au milieu rural. Plus globalement, cela renvoie à l'écosystème dans lequel les véhicules autonomes évolueront. Compte tenu de la diversité des cas d'usage, la première exigence est que le véhicule reconnaisse lui-même s'il est dans son domaine d'emploi et adapte en conséquence ses modes de délégation de conduite. Il importe donc que le véhicule autonome puisse lire la signalisation. C'est par une combinaison adéquate de la signalisation, de la connectivité et de la cartographie numérique que l'on pourra optimiser les cas d'usage du véhicule autonome. Nous avons engagé avec les acteurs concernés un travail d'identification des « amers » prioritaires.

Au 1 janvier 2016, le parc français de véhicules en circulation était estimé à près de 39 millions d'unités. Si une quarantaine d'expérimentations sont déjà en cours, il faudra vingt et un ans pour renouveler entièrement le parc automobile. ouvre, à long terme, des perspectives intéressantes en matière de sécurité routière et d'environnement, mais suscite aussi des inquiétudes en termes de sécurité et d'accessibilité. Le véhicule autonome est présenté comme un moyen radical de réduire la mortalité sur les routes et de limiter la consommation d'énergie. Dès lors que 90 % des accidents sont dus à une erreur humaine, seul le remplacement de l'ensemble du parc automobile permettra une diminution de la mortalité routière. Si, à brève échéance, la mise en service de ce type de véhicules sera réalisable sur les autoroutes, déjà dotées d'infrastructures, il n'en va pas de même pour le réseau secondaire, où se concentre l'essentiel des accidents

on circulera dans des véhicules sans chauffeur sur les autoroutes et dans les grandes villes, alors que les habitants de la ruralité seront bloqués chez eux, n'ayant plus de points sur leur permis ... Les ruraux, condamnés

Enfin, la mise en service de ce type de véhicules « sans conducteur » pose de vraies questions en matière de responsabilité en cas d'accident, mais aussi et surtout de cybersécurité. Pourra-t-on garantir aux usagers qu'ils seront protégés du piratage de leurs données personnelles ou des attaques terroristes ? La parole

Au-delà de ses conséquences directes très importantes en termes d'emplois, cette révolution aura un impact plus difficile à imaginer sur les constructeurs, dont l'activité va se transformer : on ne fabrique pas de la même manière un véhicule qui sera utilisé de 80 % à 90 % du temps

Nous devons dès aujourd'hui définir des objectifs ambitieux afin de profiter de cette révolution, et non de la subir : réduire drastiquement le nombre de véhicules individuels, diminuer la place de la voiture dans l'espace public, améliorer la qualité environnementale et la qualité de l'air,

Notre droit des assurances automobiles exclut aujourd'hui la responsabilité directe d'un objet, retenant exclusivement la responsabilité du conducteur. Or l'essor attendu de la conduite sans chauffeur pourrait multiplier les parties prenantes et introduire de nouvelles causes d'accidents, dans des conditions que le droit actuel n'appréhende pas. Qui sera responsable d'un accident mortel survenu à un croisement par temps clair,

du fabricant du logiciel, du constructeur, voire du propriétaire ? Comment assurera-t-on demain les cyberrisques liés à la possibilité de pirater des véhicules à distance ? Dans tous ces domaines, le vide juridique est total. Dans sa résolution législative du 16 février 2017, le Parlement européen propose de créer un statut juridique applicable à « tout robot qui prend des décisions autonomes ou qui interagit de façon indépendante avec des tiers Ce robot serait alors tenu de « réparer tout dommage causé à un tiers ». Faut-il plutôt retenir la responsabilité de la personne ayant programmé le robot ? Le choix sera d'autant plus complexe que de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle élaborent désormais eux-mêmes des simulations leur permettant d'apprendre dans la phase initiale, écarte le recours à un « maître d'apprentissage » et rend ainsi le critère en question obsolète avant même son adoption. Comment le Gouvernement entend-il anticiper la dimension juridique du mouvement entamé avec le véhicule sans chauffeur ? Comment permettre l'évolution de cette nouvelle économie tout en protégeant les victimes à venir

En matière de responsabilité civile, la loi Badinter de 1985 dispose que les victimes d'un accident de circulation sont indemnisées par l'assureur en responsabilité civile du véhicule. véhicule. On peut penser que cette disposition peut être transposée au cas du véhicule autonome. En revanche, en matière de responsabilité pénale, les choses sont plus complexes.

le régime permanent, il faudra tenir compte des différents cas d'usage dans lesquels coexisteront un système d'automatisation impliquant lui-même plusieurs acteurs et, selon les situations de conduite, un conducteur. Nous devons travailler avec les parties prenantes à mettre en place un cadre de responsabilité adapté, qui prenne également en compte les réflexions élaborées à l'échelon de la Commission européenne. Il devrait être présenté dans le cadre de la stratégie 2018-2020. Par ailleurs, il nous faudra concilier le besoin d'un cadre général avec la nécessité de s'adapter aux différents cas d'usage. C'est vraiment tout l'intérêt des expérimentations à venir que de permettre un dialogue avec les parties prenantes sur ces différents sujets. J'ajoute que

par dérogation, après validation par cinq instances différentes : ministère des transports, ministère de l'intérieur, gestionnaire de la voirie, autorité de la police de la circulation, autorité organisatrice des transports. Cette procédure d'autorisation des expérimentations dure en moyenne quatre mois, ce qui reste un délai important au regard des temps d'innovation très courts dans le monde du véhicule autonome. L'entreprise Valeo a ainsi été confrontée à de nombreuses difficultés pour faire rouler son véhicule autonome dans les rues de la capitale. Son objectif était de le tester sur la place de l'Étoile, réputée comme la section

Notre pays pourrait s'inspirer, par exemple, du modèle suédois Drive Me, qui consiste à faire tester cent véhicules autonomes pendant un an par des particuliers et sans ingénieur à bord.

de la cohabitation, sur les routes, des véhicules autonomes et des véhicules classiques. Réaliser des tests à grande échelle en imposant aux usagers de produire des retours d'expérience complets devrait permettre de tirer les premières conclusions. Ma question est donc simple, madame la ministre : la France est-elle prête à s'inscrire dans cette dynamique ?

avec d'autres véhicules, y compris d'autres véhicules autonomes. Toutefois, il faut maintenant passer à l'échelle supérieure, selon quatre axes. Le premier axe, c'est la mutualisation entre acteurs.

En effet, cette révolution technologique nous invite à repenser en profondeur les mobilités. Envisagé dans un cadre multimodal intelligemment conçu, le développement des véhicules autonomes est porteur de grandes promesses en matière de sécurité routière, de transition écologique et de confort de déplacement. Cependant, les questionnements et les inquiétudes écologiques, économiques, éthiques et réglementaires ne manquent pas, comme en témoigne notre débat. À dire vrai, nous n'avons à ce jour qu'une seule certitude la disparition progressive, dans les deux ou trois décennies à venir, de la quasi-totalité des emplois de chauffeur et de conducteur de taxi, de VTC, de bus, de tram, de train et de camion. Il s'agit là de près d'un million de travailleurs ! La question de leur reconversion est primordiale. Plus largement, tous secteurs confondus, ce sont de 50 % à 80 % des emplois existants qui auront disparu en 2050, selon les études qui se succèdent sur le sujet, par Il est donc indispensable de réfléchir dès maintenant à la reconversion et à l'accompagnement de ces travailleurs. De la répartition et du temps de travail à l'architecture de la protection sociale, il faut repenser toute notre organisation du travail, que ce soit autour du revenu universel ou d'autres dispositifs. L'explosion des gains de productivité nous offre une source de financement toute trouvée, que d'aucuns auraient appelée « taxe robot ». Ce n'est pas une coïncidence si ces solutions sont aujourd'hui envisagées par de grandes figures de l'économie numérique telles que Bill Gates, Mark Zuckerberg et Elon Musk, patron de Tesla, pionnier des véhicules autonomes. À nous d'anticiper ces évolutions pour transformer cette innovation en amélioration de la qualité de vie pour tous. Madame la ministre, l'inventivité technologique nous pousse à être inventifs socialement. Comment le Gouvernement envisage-t-il d'accompagner ces bouleversements ? La

Les jeunes sont particulièrement concernés, mais aussi les salariés en insertion, qui sont ainsi maintenus en situation de précarité et de fragilité. Si, dans les métropoles, les transports urbains sont une solution alternative, comment faire, actuellement, pour vivre et travailler à la campagne sans permis de conduire ? En milieu rural, l'absence de permis de conduire interdit en général l'accès à l'emploi. C'est l'un des enjeux liés au développement du véhicule autonome. Alors qu'on le présente souvent comme une menace pour l'emploi, ce qu'il est réellement pour les professionnels de la route, il pourrait aussi, paradoxalement, être un moyen d'accès à l'emploi pour des milliers de personnes, à condition que son développement s'accompagne d'une réforme du permis de conduire. Madame la ministre, pouvons-nous espérer que les véhicules autonomes de niveaux 1 à 3 pourront être conduits avec des permis spécifiques et allégés ? Le cas échéant, les véhicules de niveau 4

Parmi les chantiers à ouvrir en lien avec le développement du véhicule autonome, il y a effectivement celui du permis de conduire. Aujourd'hui, on considère que l'humain qui conduit un véhicule doit être formé, que sa formation doit avoir été validée par un examen, qu'il doit être apte à conduire, à la fois physiquement et mentalement. Pendant longtemps encore, tant qu'il s'agira de véhicules à délégation partielle, voire quasiment totale, de conduite, ces conditions devront continuer à être satisfaites. satisfaites. Même s'il existe de nombreuses fonctions d'assistance, le conducteur devra être en mesure de reprendre la main si le véhicule identifie qu'il se trouve dans un environnement qu'il ne sait pas maîtriser.

qui associera largement les professionnels automobiles, ceux de la formation, les inspecteurs du permis de conduire et la sécurité routière, ainsi que les associations, les psychologues experts de la conduite automobile. Il nous faut effectivement repenser le

ces deux domaines relevant invariablement d'un angle mort de notre réflexion. Qui peut savoir quelle sera la place de l'aérien, sous toutes ses formes, demain et après-demain ? Alors que la durée d'élaboration et de vie de nos infrastructures est particulièrement longue, nous sommes soumis à des ruptures technologiques de plus en plus brutales. Je m'interroge donc sur la place de la puissance publique dans un tel contexte, sur notre capacité collective d'anticipation, de planification et de prospective. Vous préparez une importante loi d'orientation, que vous annoncez désormais pour l'été. Comment un État stratège et svelte entend-il s'inscrire efficacement dans le temps long ? Le peut-il, madame la ministre ?

place de l'industrie ferroviaire française et de nos opérateurs dans le domaine des métros autonomes, qui sont la solution technologique de demain pour les grandes métropoles. Je puis vous l'assurer, monsieur le sénateur, la réflexion conduite au sein de mon ministère prend bien en compte l'ensemble des modes de transport,

autonome. Je l'ai dit, notre stratégie en termes de véhicules autonomes va dans le sens du développement de véhicules propres. Elle vise aussi à développer prioritairement les cas d'usage permettant de fournir de nouveaux services de mobilité

alors souligné que les enjeux techniques, économiques et stratégiques étaient planétaires. En effet, une concurrence accrue s'est mise en place entre les différents acteurs, à savoir les constructeurs traditionnels, le nouveau constructeur Tesla, les géants du numérique, comme Google, les équipementiers et toutes les firmes actives dans le domaine de l'intelligence artificielle. À titre d'exemple, le géant chinois des télécommunications Huawei travaille aussi sur le véhicule connecté. Nous constatons également que des alliances sont signées entre les différents acteurs à l'échelle mondiale. Mais, au-delà de cette dimension strictement industrielle, il y a un enjeu essentiel en matière de liberté et de sécurité.

où la collecte, la transmission et le traitement des données sont assurés par des opérateurs qui travaillent dans un contexte juridique et culturel souvent dédaigneux des conceptions européennes du respect de la vie privée.

Or la conduite sans chauffeur exigera la protection des données personnelles, car celle-ci constitue l'élément basique de la cybersécurité. Il faudra donc inventer un nouveau modèle économique : vaste programme Assurer une cybersécurité inviolable est un préalable absolu au déploiement du véhicule autonome capable d'emprunter n'importe quelle voie de circulation.

quelles mesures, notamment législatives, le Gouvernement compte-t-il prendre dans le domaine du véhicule sans chauffeur pour garantir la protection des données personnelles et un haut degré de cybersécurité ?

au travers de la loi d'orientation des mobilités, de définir un socle minimum d'informations que le propriétaire du véhicule devra recevoir sur le fonctionnement des algorithmes de délégation de conduite.

est donc nécessaire d'accompagner les innovations numériques, par l'application de préceptes ayant fait leurs preuves en matière d'architecture sécurisée, de maintien en conditions de sécurité, d'analyse de risques, de certification de sécurité adaptée aux environnements complexes. Il y a là un enjeu

On peut également saluer la décision du Gouvernement de s'emparer du sujet, en nommant un pilote de la stratégie nationale sur les véhicules autonomes, à savoir Anne-Marie Idrac. Pourtant, le risque de voir nos champions nationaux distancés par les industriels étrangers est bien réel

peuvent faire librement évoluer leur législation afin que celle-ci ne soit pas un obstacle à l'évolution technologique. Les États-Unis ne se sont d'ailleurs pas privés de le faire en septembre dernier, en votant un texte permettant la circulation, à titre expérimental, de 100 000 véhicules autonomes sur toutes les voies du pays. Quant à la Chine et au Royaume-Uni, ils ont signé en novembre dernier un accord de coopération sur la conduite intelligente. Très clairement, l'article 8 de la convention de Vienne bride dangereusement nos industries. Aussi, madame la ministre, pouvez-vous nous dire comment le Gouvernement entend faire sauter des verrous qui pourraient s'avérer très rapidement préjudiciables au maintien de nos champions nationaux dans cette course technologique et comment il peut oeuvrer pour que notre droit s'adapte à ces mutations ? La parole est à Mme la ministre.

l'intégration des dispositifs d'aide ou d'assistance à la conduite, l'interprétation que l'on peut en avoir étant qu'il permet de couvrir jusqu'aux niveaux 3 et 4 d'automatisation. En 2017, nous avons mis sur la table une réglementation horizontale visant à adapter l'un des règlements afin de permettre de traiter tous les cas d'usage et de prévoir que les exigences soient proportionnées et spécifiques aux risques.

l'autopilote du véhicule Tesla accidenté, ébloui par une forte luminosité, n'avait pas repéré la remorque d'un camion ... Pour remédier à ce problème, et comme l'a très bien souligné notre collègue Pierre Médevielle, coauteur du rapport de la commission des affaires européennes, nous devrons faire évoluer nos équipements routiers. Il pourrait être question de créer de nouveaux marquages au sol ou de permettre aux panneaux de signalisation d'émettre des signaux radio à destination des usagers connectés. Mais, bien entendu, tout cela un coût

les enjeux, d'identifier les cas dans lesquels il peut être intéressant d'équiper plus lourdement l'infrastructure et ceux dans lesquels le véhicule devra se débrouiller seul,

Les réseaux de communications électroniques seront en effet indispensables au fonctionnement des véhicules autonomes, dont nous savons qu'ils tiendront une place essentielle dans les offres futures de mobilité et constitueront un atout dans la lutte contre l'insécurité routière. Dans ce contexte, notre pays doit se doter rapidement d'un cadre réglementaire, afin que les constructeurs automobiles et les différents acteurs puissent continuer à travailler au développement du véhicule de demain dans des conditions satisfaisantes et adaptées, que la gouvernance des déploiements soit définie

entre le véhicule et l'infrastructure. Il s'agit d'une expérimentation à grande échelle, qui associe de multiples acteurs : collectivités locales, gestionnaires routiers, constructeurs automobiles- en l'occurrence PSA et Renault -, universités, centres de recherche, opérateurs de téléphonie, fournisseurs de services de sécurité. Ce projet vise à déployer 3 000 véhicules sur 2 000 kilomètres de routes, répartis entre cinq sites- l'Île-de-France, l'autoroute A4, l'Isère, la rocade de Bordeaux et la Bretagne

les capacités financières sont colossales, avec Fiat est préoccupant, Google s'arrogeant le domaine de l'intelligence artificielle. Partagez-vous cette préoccupation ? La rupture à laquelle nous allons assister sera tout autant technique que culturelle ou juridique, ce

Alors que le Gouvernement prépare un projet de loi visant à élaborer un cadre législatif renouvelé pour les transports, je tiens, madame la ministre, à vous interroger sur vos intentions concernant les véhicules autonomes. Le développement d'une conduite automatisée et sécurisée est de nature à permettre l'émergence de nouvelles formes de mobilité, à la frontière entre véhicules individuels et transports collectifs.

Par ailleurs, les enjeux industriels et les conséquences sur l'emploi sont majeurs. L'industrie automobile emploie plus de 440 000 salariés en France la capacité de notre pays à accompagner ses développements est cruciale à l'heure où des acteurs de rang mondial investissent massivement le secteur, avec l'appui des États-Unis ou de l'Allemagne, par exemple. Je souhaiterais donc connaître les intentions précises du Gouvernement en la matière, en particulier les mesures législatives qu'il envisage de faire adopter pour permettre le développement plus rapide des véhicules autonomes en vue de faire de la France un pays de cette technologie d'avenir.

il faudra décourager l'« autosolisme » ou, en tout cas, encourager le partage, que ce soit par la création de voies dédiées ou par le développement de zones à circulation restreinte,

une priorité, que l'État soutiendra. Plus généralement, je souhaite accompagner le déploiement des solutions de nouvelle mobilité dans les territoires peu denses

voilà encore quelques années, le véhicule autonome était encore un concept très éloigné de notre quotidien, les choses se sont beaucoup accélérées depuis : désormais, le véhicule autonome est une réalité. Une nouvelle solution de mobilité arrive sur nos routes et dans nos villes, une innovation majeure qui va engendrer de grands changements dans la société, mais aussi dans l'industrie. L'enjeu pour la France est donc crucial. L'État doit tout mettre en oeuvre pour que nous ne manquions pas ce rendez-vous, qui constitue une véritable chance sur les plans économique et social. En effet, la France regorge de talents, de formations de qualité, de savoir-faire reconnus qui doivent nous permettre de développer les meilleurs systèmes d'autonomie au monde. de ces enjeux, qui sont aussi ceux de la révolution des transports et de la réorganisation des zones urbaines, il est nécessaire que l'État puisse structurer et coordonner l'ensemble de la filière- constructeurs, équipementiers, professionnels du numérique -pour définir une stratégie globale de développement. Au vu de ce qui se passe à l'échelle mondiale, force est de constater que nous sommes à la peine. Faute d'un cadre d'expérimentation volontariste et ambitieux, et du fait d'une réglementation très contraignante, nous pourrions manquer ce rendez-vous. La circulation automobile n'est pas régie par le droit de l'Union européenne et chaque État membre garde la main sur les autorisations d'expérimentation sur son propre sol. Actuellement, les concepteurs doivent transmettre un dossier d'autorisation à la Direction générale de l'énergie et du climat, qui doit ensuite être validé par le ministère des transports, celui de l'intérieur, l'autorité de police, le gestionnaire de la voirie et, enfin, l'autorité organisatrice des transports Ce cadre juridique constitue un frein au développement de l'intelligence artificielle, et donc du véhicule autonome, puisqu'au lieu d'accompagner ce mouvement, il le ralentit. C'est pourquoi

l'intégration des véhicules autonomes dans un système global de mobilité en encourageant les usages partagés et en renforçant le rôle des autorités organisatrices de la mobilité. Il faut améliorer la structuration de nos expérimentations pour préparer la future réglementation technique,